reprise. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

santé publique. Nous souhaitons que les parlementaires soient représentés au sein de cet observatoire, de manière à lui garantir une impulsion politique. D'une part, cette disposition contribuera à la diffusion de l'information auprès de nos concitoyens et à la sensibilisation des Français à un enjeu majeur de santé publique qui touche l'ensemble de la population, en premier lieu nos enfants. En effet, la pollution de l'air intérieur représente un risque un risque pour 95 % des enfants et 5 % des foetus. Ces chiffres témoignent de la nécessité de donner une impulsion politique à cet organe afin d'en accroître la visibilité. D'autre part, cet amendement s'inscrit dans la logique de la proposition de loi récemment adoptée visant à garantir la présence des parlementaires dans les organismes extraparlementaires. Cette représentation au sein de l'observatoire permettra en effet de favoriser les nécessaires débats de fond au sein des chambres parlementaires sur un sujet qui, par sa nature et son importance, peut représenter une source d'inquiétude légitime pour nos concitoyens.

Mme Jacky Deromedi. L'article 21 E donne expressément compétence au préfet, dans les zones couvertes par un plan de protection de l'atmosphère, pour interdire l'usage d'appareils de chauffage polluants, en particulier les foyers ouverts et, potentiellement, les appareils de chauffage au charbon. Or les dispositions actuelles de l'article L. 222-6 du code de l'environnement confèrent déjà une base juridique à la prise de telles mesures, en donnant la possibilité à l'autorité compétente de prendre les mesures préventives, d'application temporaire ou permanente, destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique. Cet amendement vise donc à supprimer l'article 21 E du projet de loi. Quel est l'avis de la commission ? La commission

: La parole est à Mme Josiane Costes. Le contrat de vente d'immeuble à rénover est peu usité en raison du cumul en une seule et même personne des responsabilités de vendeur et de maître d'ouvrage des travaux de rénovation. Afin de développer davantage les ventes d'immeubles accompagnées de travaux de rénovation, le présent amendement a pour objet de créer un nouvel outil contractuel, à savoir un contrat de promotion-rénovation pouvant être conclu concomitamment à tout contrat de vente d'un logement, avec une personne autre que le vendeur. Celle-ci fera procéder aux travaux de rénovation en se chargeant des opérations juridiques, administratives et financières correspondantes. Nous prévoyons également que les contrats de vente et de promotion-rénovation devront être précédés obligatoirement d'une promesse unique engageant le vendeur, l'acquéreur et le promoteur-rénovateur. de cet amendement proposent de créer un contrat intermédiaire, le contrat de promotion-rénovation, entre la promotion immobilière et la vente d'immeuble à rénover.

L'article L. 111-3-2 a été intégré dans le code de la construction et de l'habitation en vue de protéger les entreprises artisanales qui exécutent des marchés en groupement momentané d'entreprises. Il est ainsi prévu, notamment, de faire figurer dans les marchés de moins de 100 000 euros les mentions expresses de l'existence ou non de la solidarité des cotraitants envers le maître d'ouvrage, ainsi que du nom et de la mission du mandataire commun des cotraitants.

En effet, il a créé la possibilité, pour les maîtres d'ouvrage, de soulever des vices de pure forme susceptibles d'entraîner la nullité du marché. La nullité peut, ainsi, être invoquée à tout moment : juste après la signature du marché, en cours d'exécution ou bien encore juste avant sa réception. Les conséquences pour les entreprises sont désastreuses : les dispositions contractuelles ne peuvent plus être invoquées, car elles sont toutes caduques. Ainsi, le prix du contrat peut, en particulier, être réétudié. Aussi certains maîtres d'ouvrage utilisent-ils cette arme pour obtenir la nullité du marché afin de revoir à la baisse le prix du marché et de pratiquer des offres anormalement basses. Le vice de forme a, par effet d'aubaine, des conséquences sur le fond du contrat. du contrat. La sanction en l'absence des mentions prescrites par l'article L. 111-3-2 du code de la construction et de l'habitation est disproportionnée par rapport au manquement,

? La commission est défavorable à ces amendements, qui tendent à établir, par principe, l'absence de solidarité entre les cotraitants dans un marché privé de cotraitance. Là encore, sans retour de terrain suffisant et sans évaluation précise

la délégation sénatoriale aux outre-mer a réalisé en 2016 un rapport d'information relatif à la situation du secteur du bâtiment et des travaux publics au regard des normes techniques.

En effet, si l'existence de surprimes est largement liée à la prégnance des risques naturels dans ces territoires, une évaluation claire du différentiel et une analyse précise de ses justifications semblent nécessaires si l'on souhaite mieux maîtriser ces coûts.

interpellés par les élus locaux au sujet de leurs très grandes difficultés à faire sanctionner les infractions au permis de construire ou au code de l'urbanisme, c'est-à-dire les constructions sans permis.

y a une certaine réserve de la part de la magistrature judiciaire et du parquet à entrer dans l'analyse de la bonne application de textes d'urbanisme, qui relèvent du droit administratif.

comme je le souhaite, un chapitre particulier de sanctions administratives qui s'ajouteraient aux sanctions pénales du code de l'urbanisme. Nous pourrions l'introduire, si les délais le permettent, au travers du projet de loi sur la justice. Quel est l'avis de la commission ? ? Pour intéressante et légitime que soit votre proposition, monsieur Richard, elle contredirait l'application de la prescription de dix ans, et le nouveau propriétaire d'un bien pourrait se retrouver dans l'obligation de procéder à la mise en conformité, alors qu'il n'est pas responsable de la non-conformité.

Cet amendement soulève une question pertinente. Pour autant, l'acquéreur n'a pas à mentionner, dans le contrat de vente, l'usage qu'il entend faire du bien. Il semble donc juridiquement difficile de prévoir un régime spécifique d'information de l'acquéreur lorsque celui-ci souhaiterait démolir

24 opère une réforme d'ampleur du contentieux de l'urbanisme. Nous le savons tous, pour l'avoir régulièrement éprouvé dans l'exercice de nos mandats locaux, les recours abusifs sont devenus des armes utilisées par certains dans le seul but de ralentir des opérations.

Rappelons que la notion de recours abusif, introduite par la loi Duflot, visait explicitement les manoeuvres frauduleuses et le chantage par le biais de recours crapuleux.

de cette présomption. Seules celles qui exercent leur activité depuis trois ans au moins, qui sont régulièrement déclarées et agréées par l'autorité administrative, sont concernées. Ces précautions étant prises, il est de bon sens de considérer que les associations de protection de l'environnement ne sont pas là pour faire chanter les promoteurs immobiliers au moyen des recours abusifs. Laissons la justice décider du bien-fondé des recours intentés. Cette présomption est donc indispensable pour éviter que,, les grandes entreprises du BTP tentent de faire tomber des recours en les faisant passer pour des recours abusifs. abusifs. Cela alourdirait la procédure judiciaire. Considérant les moyens financiers respectifs des parties prenantes, cet alourdissement de la procédure ne peut être qu'au détriment des associations. Cette présomption équilibre le rapport de force entre les associations et les grandes entreprises. Elle permet de ne pas dissuader des associations d'intenter une action en justice

L'ordonnance, adoptée par le conseil des ministres du 17 juillet 2013, relative au contentieux de l'urbanisme, dite « ordonnance Duflot », si elle a pour objectif de lutter contre les recours manifestement malveillants, prévoit que les associations de protection de l'environnement bénéficient, compte tenu de leur objet, d'un régime de protection particulier fondé sur la présomption que leurs recours obéissent, par principe, à un motif d'intérêt général. En pratique, on constate que des associations forment des recours dilatoires et abusifs contre des projets de construction ou d'aménagement qui n'ont aucune incidence sur les intérêts qu'elles se sont donnés pour objet statutaire de défendre et de protéger. La seule circonstance que ces associations soient régulièrement déclarées et qu'elles aient pour objet principal la protection de l'environnement les protège de tout risque de condamnation à des dommages et intérêts prononcée par le juge administratif sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. L'immunité dont ces associations bénéficient les encourage à contester de manière systématique certains projets de construction et d'aménagement. Afin de lutter contre ce type de recours abusifs, il serait utile de supprimer cette immunité, et donc de modifier l'article du projet de loi en insistant sur l'obligation que le recours soit en rapport direct avec l'objet statutaire de l'association. Il s'agit non pas de limiter les recours introduits par les associations pour assurer la défense de leurs intérêts statutaires, mais de combattre les recours formés par des associations

résulte très clairement des dispositions de l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme et de l'article 635 du code général des impôts qu'une transaction prévoyant, en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature, le désistement du recours en annulation formé contre une autorisation d'urbanisme, doit, à peine de nullité de cette contrepartie, faire l'objet d'un enregistrement auprès des services fiscaux dans le mois suivant la signature du protocole transactionnel. La sanction d'un défaut d'enregistrement de la transaction dans ce délai d'un mois est donc la nullité de la contrepartie offerte par le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme au requérant qui a accepté de se désister. Certes, l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme ne mentionne pas expressément que les contreparties enregistrées tardivement sont sans cause, mais cette sanction est induite par les dispositions mêmes de cet article. En effet, le premier alinéa de l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme pose le principe

La circonstance que l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme ne prévoit pas expressément que, faute d'un enregistrement de la convention dans un délai d'un mois, la contrepartie prévue par une transaction est nulle, a conduit certains tribunaux à ne pas sanctionner de nullité la contrepartie prévue par une transaction enregistrée au-delà du délai d'un mois. La rédaction de l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme n'est donc pas satisfaisante, dans la mesure où la sanction d'un défaut d'enregistrement de la convention au-delà du délai d'un mois ne résulte pas du texte même de cet article, contrairement à ce que le rapporteur du projet de loi ÉLAN à l'Assemblée nationale a affirmé pour demander le retrait de l'amendement déposé par le député Jacques Cattin. La position adoptée par ce rapporteur va à l'encontre de l'objectif des auteurs de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme : lutter contre les recours abusifs en matière d'autorisations d'urbanisme. Par cet amendement, nous entendons donc clarifier l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme.

et de sécuriser le pétitionnaire dans son acte de construire. Nous proposons donc, au travers de cet amendement, qu'à compter de l'enregistrement de la requête introductive d'instance le tribunal administratif délivre un calendrier de procédure permettant d'avoir une meilleure connaissance de la date de l'audience. Quel

amendement vise à exclure l'engagement de la responsabilité pénale du bénéficiaire d'une autorisation de construire qui, de bonne foi, engage les travaux. Cela s'inscrit dans un cas où l'autorisation de construire est déjà définitive,

avec un certain manque de prudence

Monsieur le ministre,

le paiement des impositions afférentes à cette autorisation est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle devenue définitive ». Je vous demande

en 2013. L'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, qui avait prorogé pour un an un dispositif permettant d'améliorer les contentieux en matière d'urbanisme.

rechercher un accord entre l'autorité compétente pour élaborer les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, ou les cartes communales, et les autres personnes associées à cette

Nous en arrivons à un article sensible de ce projet de loi, celui qui organise les regroupements d'organismes d'HLM. Nous sommes face à une volonté cohérente et généralisée d'aller vers la constitution de structures géantes, partout sur le territoire, et ce en dépit des exigences de proximité. Ces mégastructures seront déconnectées des besoins des territoires et des habitants. Après le regroupement à marche forcée des intercommunalités, voici donc le regroupement à marche forcée des organismes d'HLM.

de très petits offices très performants et de très gros offices complètement déconnectés des besoins. En revanche, le lien territorial de proximité est essentiel pour garantir l'humanité du traitement des demandes. Nous restons pour notre part opposés, quel que soit le seuil défini, à ces mariages forcés qui n'augurent rien de bon pour les locataires ou pour l'aménagement du territoire. Le seul enjeu est bien celui de la mutualisation des fonds propres et des moyens de faire remonter cet argent.

comment donner au secteur HLM de nouvelles marges de manoeuvre par des aides à la pierre renforcées, par un recentrage sur ses missions essentielles. À l'inverse, vous engagez une course folle au gigantisme. Nous demanderons donc la suppression de cet article. La parole est à M. Fabien Gay,

L'organisme créé sera alors le seul à pouvoir prétendre aux prêts bonifiés de la Caisse des dépôts et consignations. En procédant de la sorte, le Gouvernement favorise une centralisation qui risque de nuire à la proximité et au lien avec les territoires. au-delà des seuils fixés, une telle démarche n'a pas les mêmes conséquences en tout point du territoire. Le nouvel organisme pourra couvrir des territoires très différents, qui présentent de véritables spécificités. Les mariages forcés engendrent rarement des relations harmonieuses ! Sans réel projet de territoire qui motiverait une fusion, le risque est de perdre en efficacité, à rebours À la place de ces regroupements obligatoires, nous proposons des rapprochements sur la base du volontariat, qui s'opéreraient en raison de réelles similitudes, de réels besoins ou de projets coconstruits. Ces rapprochements forcés risquent également de créer de véritables usines à gaz et de causer une déconnexion des besoins de proximité, d'une rupture avec Or, derrière la question des logements sociaux, il y a bien évidemment cette dimension humaine, et parfois des situations de grande précarité. Pour certains, se rendre à un rendez-vous au siège du nouvel organisme

Nous ne souhaitons pas qu'une organisation proche des territoires, garante d'un certain équilibre et d'une proximité, disparaisse au bénéfice d'une recherche de profit ou de rationalisation par la fixation de seuils arbitraires, sans lien avec nos territoires. La parole

que d'expliquer que l'on va réussir, en regroupant les organismes d'HLM, à « rationaliser » l'utilisation de l'argent dédié au logement social. Il faut dire que, à Bercy, ils aiment bien ce qui leur ressemble, comme si jamais ils ne s'étaient trompés

pour 4,3 millions de logements. En Allemagne, il y a 3 000 bailleurs sociaux, soit quatre fois plus, pour 6 millions de logements, une fois et demie plus.

la restructuration, étalée sur trois ans, des organismes de logement social donnera demain à ces derniers la possibilité de se rassembler pour agir avec plus d'efficacité.

Bien au contraire, mes chers collègues, ce projet de loi a été conçu de manière à atteindre un bon équilibre entre la nécessaire proximité et la mutualisation. Ainsi, un organisme locatif social qui n'aurait pas une taille suffisante, mais qui serait situé dans un territoire où les bailleurs sont peu nombreux et le parc réduit, ne serait en aucun cas soumis à l'obligation de regroupement.

de l'efficacité de la gestion, de la production et de la rénovation de logements sociaux représente un devoir moral de l'État à l'égard des citoyens, notamment des plus modestes d'entre eux,

La commission a beaucoup travaillé pour aller dans le sens des regroupements et essayer de trouver des solutions. On ne va pas refaire le débat sur le volet budgétaire. Notre ambition était à la fois de

Vous avez dû accepter, Mme la rapporteur l'a dit, des réductions drastiques du budget du logement, comme jamais on en avait vu depuis des années, quels que soient les gouvernements qui se sont succédé.

Vous ne parlez pas des élus locaux. Depuis des années, des relations de confiance, parfois conflictuelles, se sont développées entre des offices d'HLM ou des SA d'HLM et des élus locaux. D'ailleurs, les élus locaux ont apporté des garanties au logement social.

le secrétaire d'État, sans doute est-ce parce que je n'appartiens pas au nouveau monde, mais il y a un élément de logique que j'ai du mal à comprendre dans l'attitude du Gouvernement. Alors que vous proposez d'inscrire dans la Constitution un droit à la différenciation,

de la construction de logements dans les zones très urbanisées et le délaissement des zones rurales et des zones les plus excentrées. J'appelle donc le Gouvernement à bien réfléchir avant de mettre en oeuvre des dispositions d'ordre général, qui auraient des conséquences particulièrement négatives.

C'est une position qui a été défendue à l'Assemblée nationale et qui emporte également l'adhésion ici de la majorité du Sénat. Mais le Gouvernement tient à un seuil et, nous l'avons compris, vous ne reculerez pas, La commission a abaissé le seuil à 10 000 logements, au lieu de 15 000 logements. Nous sommes satisfaits de cette première évolution, car nous sommes nombreux à le dire : la taille ne présume en rien de l'efficacité de la gestion d'un organisme. Plutôt que la taille d'un organisme, c'est la concentration géographique de son patrimoine qui constitue l'élément prépondérant de la maîtrise des coûts de gestion. Cet amendement vise à proposer une deuxième évolution évolution : confier aux comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement, les CRHH, une mission de pilotage et d'évaluation des projets de regroupements, pour assurer la pertinence financière de ces derniers et la capacité des organismes à rester connectés avec les territoires. Le CRHH pourra aussi, le cas échéant, proposer au préfet de région une modulation du seuil des 10 000 logements pour tenir compte des spécificités de l'offre et de la demande de logements sociaux sur le territoire concerné.

ESH, ils pourraient appartenir à la fois un groupe et à une SAC. Par principe d'équité et d'égalité entre organismes de logements sociaux,

de l'efficacité qu'attendent les collectivités locales, et encore plus les habitants, des organismes de logements sociaux. L'organisme doublement rattaché risque très vite de se trouver pris dans des contradictions insolubles. En cas de contradiction, quelle politique l'organisme devra-t-il privilégier ? Une double appartenance sera pour nous, me semble-t-il, source de complexité

d'une démarche prônant la concertation et afin d'améliorer la démocratie participative, nous souhaitons, tout simplement, renforcer le rôle des représentants des locataires au sein des bailleurs. Il convient de les associer et de les consulter pendant les phases d'élaboration du cadre stratégique patrimonial. dans les missions du cadre stratégique patrimonial de permettre aux organismes de réfléchir à l'attractivité de leur patrimoine, en fonction de la connaissance des marchés locaux de l'habitat et des attentes des locataires comme des demandeurs de logement, cela ne peut se faire qu'à l'approbation de la majorité des représentants des locataires. Il paraît aujourd'hui indispensable que des décisions de cette importance soient prises en écoutant les premiers concernés. Nous pouvons tous être d'accord pour dire que les choix d'investissement et de gestion d'un parc auront des conséquences directes sur la vie de ses locataires : ils ne peuvent donc se faire sans l'accord de leurs représentants. Quel est l'avis de la commission ?

des engagements en matière d'accès au logement pour les personnes à mobilité réduite, en situation de handicap ou en perte d'autonomie, en précisant que ceux-ci doivent être pris en compte dans le cadre de l'élaboration de la CUS. Considérant que cet amendement est satisfait,

L'objet des sociétés de coordination prévoit de multiples prérogatives et mesures visant à encadrer et contrôler les activités et moyens d'organisation des organismes qui détiennent son capital. Il ne paraît pas nécessaire d'imposer, en outre, une représentation des membres de la SAC au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Il appartiendra aux actionnaires d'en décider lors de la constitution de la société de coordination et d'en préciser les modalités au travers des clauses des statuts. Le présent amendement vise donc à permettre, pour les SAC qui le souhaitent, de faciliter l'échange d'informations entre elles et les organismes qui la composent. Quel est l'avis de la commission ?

Nous proposons de supprimer l'alinéa 40 de l'article 25, qui prévoit que les sociétés de coordination appellent des cotisations auprès de leurs membres pour l'accomplissement de leurs missions. Le projet de loi prévoit déjà que les « groupes d'organismes de logement social peuvent facturer des redevances ou des cotisations aux associés ou membres du groupe en contrepartie des avantages procurés En outre, le terme « cotisation » ne paraît pas adapté à une société et laisse entendre que les SAC seraient rémunérées, pour les services rendus à leurs membres, uniquement par une cotisation globale, et non par des facturations correspondant à la nature à la nature du service rendu. Un tel système est susceptible de poser des difficultés, sur le plan tant comptable que fiscal : comment distinguer, au sein d'une cotisation globale, la part qui correspond à des activités relevant du service d'intérêt économique général de celle qui correspond à d'autres activités Cette difficulté risquerait de conduire à une fiscalisation globale de ces cotisations, alors que certaines prestations rendues par la SAC peuvent être exonérées de TVA et d'impôt sur les sociétés.

Les mesures que les SAC peuvent décider pour garantir la soutenabilité financière du groupe et de chacun des organismes qui le constituent

contribue au rétablissement financier des bailleurs sociaux en difficulté ou en situation de fragilité et participe à l'ingénierie des projets de renouvellement urbain. Sur ce dernier point, il ne faut pas oublier que de nombreux organismes ont pu ainsi assumer de très importants investissements, utiles aux quartiers, et ce dans un délai extrêmement raccourci. Il est donc essentiel, pour les organismes d'HLM, même regroupés en SAC,

amendement vise à améliorer la rédaction relative à l'établissement des comptes combinés par la société de coordination. Les comptes combinés sont élaborés non par la société, mais par l'expert-comptable. Ils sont établis et publiés par la société, qui combine ses comptes avec ceux de ses actionnaires organismes de logements sociaux. Quel est l'avis du Gouvernement ?

En l'état actuel du projet de loi, deux compétences optionnelles des SAC sont réservées aux organismes d'HLM : la prestation de services de la SAC pour le compte de ses actionnaires dans toutes les interventions de ces derniers sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu'ils gèrent ; la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction neuve, rénovation ou réhabilitation d'ensembles immobiliers par la SAC pour le compte de ses actionnaires. Or les SEM agréées en application de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, qui sont également parties prenantes de ces nouvelles sociétés, ne sont pas visées par le texte actuel.

de ces derniers sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu'ils gèrent ; la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction neuve, rénovation ou réhabilitation d'ensembles immobiliers par la SAC pour le compte de ses actionnaires.

-d'être présentes jusqu'à hauteur de 50 % du capital des sociétés anonymes de coordination. Cette disposition permet d'offrir aux élus une réponse globale, dont ils sont de plus en plus demandeurs pour leurs territoires en matière d'habitat, en autorisant l'ensemble des EPL intervenant dans ce domaine par des activités relevant

des SAC, qui doivent rester spécialisées dans le logement social, et risquent, à terme, de conduire à une remise en cause du statut HLM de cette structure. Une telle faculté accordée aux SEM non agréées

sociaux est une solution rigide, qui expose par principe à la méconnaissance des situations particulières ou des situations futures que l'on n'aurait pas pu prévoir. Absolument ! Si les circonstances locales évoluent, il faut donc revoir la loi.

après avis conforme du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, en tenant compte des spécificités de l'offre et de la demande de logements sociaux sur le territoire. Cette solution me semble beaucoup plus souple et adaptée aux réalités locales. L'amendement

Un tiers des organismes seraient donc exemptés de cette obligation de regroupement et ne pourraient donc constituer l'ossature des futures sociétés de coordination territoriale. Le présent amendement vise par conséquent à adopter une solution intermédiaire, en fixant les seuils à 12 000 logements et 40 millions d'euros de chiffre d'affaires.

de région, sur avis des comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement, de moduler par arrêté le seuil des 10 000 logements sociaux. Il s'agit d'adapter la taille des regroupements, pour tenir compte des spécificités locales de l'offre et de la demande de logements sociaux, et de rester connecté avec les territoires concernés.

de certaines agglomérations qui présentent des caractéristiques très particulières, comme celles des territoires de montagne qui accueillent des travailleurs saisonniers. Il a donc pour objet de permettre des dérogations en matière de logement social en abaissant le seuil.

? L'amendement n° 377 rectifié vise à supprimer toute fixation d'un seuil dans la loi et à renvoyer la définition du seuil

le ministre, nous sommes très nombreux à demander qu'il n'y ait pas d'effet couperet. Vous aviez fait des ouvertures en ce sens à l'Assemblée nationale en vue de la navette parlementaire. La discussion sur le point d'équilibre à trouver pour adapter la taille des regroupements

Elle a été supprimée en commission, au motif qu'un seul territoire était concerné. Nous estimons pourtant que ce rattachement dérogatoire était justifié par des raisons de cohérence territoriale-

de taille significative, mais qui n'atteignent pas immédiatement la taille des 10 000 logements. Par ailleurs, cette dérogation est réservée à des territoires comportant plus de cinq OPH. Obliger ces derniers à constituer un groupement en sus d'une fusion, significativement lourde en termes de coûts et de délais compte tenu du nombre d'OPH concernés, nuirait durablement à la capacité de ces derniers à remplir leur mission première, à savoir loger, construire

vous proposez d'exonérer de l'obligation de regroupement les OPH ayant dû fusionner en application de l'article 28 du projet de loi. La commission a supprimé l'exonération à laquelle vous faites référence, qui ne concernait qu'un seul EPT. Elle émet donc, par cohérence,

de respecter ces deux obligations. Je pense que c'est la bonne formule- elle correspond d'ailleurs à la demande des organismes qui sont visés par ces deux dispositifs.

tous les acteurs dans un même organisme indépendamment de leur forme juridique présente des risques pour l'intérêt général. Ne pas tenir compte de leurs spécificités pourrait aboutir, si on les oblige à se regrouper dans des structures encore mal définies, à privatiser totalement le logement social de proximité, oubliant que les offices ont été constitués avec l'argent des locataires les plus modestes, que les emprunts ont été garantis par les collectivités de référence, c'est-à-dire les communes, sans compter l'ampleur des subventions versées par les collectivités publiques partenaires. Il est donc proposé ici de créer une dérogation au seuil de regroupement, dans le cas où les offices publics auraient déjà tous fusionné ou s'il n'en restait qu'un seul sur le territoire. Quel est l'avis de la commission ?

en deçà duquel les organismes d'habitations à loyer modéré ont l'obligation d'appartenir à un groupe, tel que le définit l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation. Des exceptions ont néanmoins été prévues aux alinéas 52 à 54 de l'article 25, s'agissant des organismes qui sont seuls à avoir leur siège dans un département, ou dont l'accession sociale à la propriété représente l'activité principale. Comme tout seuil, ce chiffre de 10 000 logements ne tient pas compte d'éventuelles spécificités locales et risque d'abîmer certaines dynamiques territoriales. La prise en compte de la réalité de nos territoires est un enjeu essentiel des politiques d'aménagement. Or un seuil national unique nous apparaît ne pas répondre à cet objectif. La dérogation que le présent amendement, dérogation accordée par l'État le préfet du département dans lequel l'organisme a son siège, après avis du conseil départemental et du conseil régional, est de nature à prendre en compte la réalité des situations locales, sans contrevenir de manière visible aux objectifs de la loi.

toujours pas quand cette réforme sera engagée. En tout cas, on ne peut pas nous demander de nous organiser selon une logique territoriale dont on ne sait pas ce qu'elle sera dans six mois, dans un an ou dans deux ans. Puisque la réforme du Grand Paris n'est pas encore prête,

Il me semble que les conditions de retrait de l'agrément sont très encadrées. Il me paraît important que les sociétés d'économie mixte soient placées, de ce point de vue, dans les mêmes conditions que les organismes d'HLM, en ayant une activité minimale.

minoritaires. Or il n'y a que deux manières de consolider les chiffres d'affaires des sociétés dans lesquelles on détient des participations. Soit en compte au prorata de la détention du capital, soit on compte à 100 %, uniquement les sociétés dans lesquelles on détient des participations majoritaires. C'est cette dernière solution qui est retenue, par cohérence avec la définition des groupes d'organismes de logement social. Monsieur le sénateur, votre proposition consiste en réalité à compter 100 % des chiffres d'affaires pour tous les actionnaires, ce qui entraînerait des doubles comptes

de 2021 à 2026. On parle souvent de l'instabilité de la loi comme d'un problème pour les acteurs économiques et pour les acteurs du logement en particulier.

l'amendement n° 561. Les organismes de logement social viennent de mettre en place la réduction de loyer de solidarité. Ils doivent en tirer les conséquences. Ils vont ainsi devoir s'occuper de la vente de logements, revoir leurs conventions le niveau de production de logements sociaux, trouver les niveaux pertinents de regroupement, et intégrer l'ensemble des réformes prévues par le projet de loi, le tout dans un contexte électoral que vous connaissez tous et qui, d'ici à 2020, est peu propice à mener efficacement les réformes. Notre amendement a pour objet de décaler la mise en oeuvre des regroupements d'une année, au 1janvier 2022,

Cette situation durera seulement le temps que les partenaires acquièrent une partie du capital de la SA HLM, permettant de ramener l'importance des participations des collectivités à un niveau n'excédant pas les deux tiers du capital. Il s'agit donc d'une disposition transitoire.